Monsieur le président, je souhaite procéder à plusieurs rectifications de votes sur le projet de loi portant création de l'Office français de la biodiversité et de la chasse, modifiant les

débat nous est apparu d'autant plus nécessaire que le programme de stabilité présente cette année une double particularité. D'une part, il est l'occasion pour le Gouvernement de mettre à jour la trajectoire au regard des mesures adoptées fin décembre, dans un contexte particulier dont nous nous souvenons tous de répondre aux préoccupations exprimées par le mouvement sur les ronds-points. D'autre part, la programmation pluriannuelle a été établie indépendamment des conclusions tirées par le Président de la République du grand débat national, alors même qu'elles risquent fort d'avoir un impact non négligeable sur la trajectoire budgétaire.

Pour 2019 et 2020, la révision à la baisse des perspectives tient essentiellement à un « effet base » défavorable et au ralentissement du commerce et de l'économie européenne qui pèse sur les exportations françaises. En revanche, la demande intérieure resterait dynamique. Le scénario de moyen terme, pour 2021 et 2022, est également revu à la baisse, ce qui constitue une première depuis le début du quinquennat. Le Gouvernement ne retient plus l'hypothèse que l'économie française entrerait dans une phase de légère « surchauffe » en fin de quinquennat.

un. Or il s'agit d'une situation atypique. Pour la suite du quinquennat, le Gouvernement retient l'hypothèse raisonnable d'un retour à une élasticité unitaire. S'agissant de la remontée des taux d'intérêt, le Gouvernement continue à faire l'hypothèse d'une remontée au rythme de 75 points de base par an, centrale européenne, la BCE, de ralentir la normalisation de sa politique monétaire. Il s'agit d'un scénario particulièrement conservateur. Certes, la prudence peut se justifier,

Venons-en maintenant au sujet qui nous intéresse principalement : la trajectoire budgétaire retenue par le Gouvernement. Je le dis, le nouveau scénario proposé apparaît particulièrement dégradé. Certes, d'un côté, l'exécution 2018 a été légèrement plus favorable qu'escompté, permettant ainsi au Gouvernement de disposer d'un « effet base » positif de 0,1 point. Mais, de l'autre côté, la dégradation des perspectives de croissance de 2019 à 2022

la réduction de la part des prélèvements obligatoires dans le PIB devrait quant à elle être plus importante qu'escompté, mais, à l'issue du quinquennat, rappelons-le, le poids de ces prélèvements resterait néanmoins supérieur de 1,7 point à celui qui était observé avant la crise financière. Le quinquennat de M. Macron permettra juste d'effacer les excès du quinquennat de M. Hollande. Alors, que penser de cette nouvelle trajectoire budgétaire ? Il convenait indéniablement de répondre à la crise communément appelée des « gilets jaunes » et, par-delà, aux attentes des Français.

Lors de la gestion de la crise financière, la France a choisi un redressement plus progressif- c'est le moins que l'on puisse dire - de ses comptes publics, afin de ne pas fragiliser la timide reprise économique. Si cette stratégie budgétaire peut se comprendre, sa crédibilité repose néanmoins

actuel paraît doublement favorable. D'une part, l'écart de production est pratiquement résorbé à l'issue de l'exercice 2019 et devrait même être positif à compter de 2020 ; d'autre part, la France bénéficie depuis 2017 d'un effet « boule de neige » positif, qui facilite la réduction du ratio d'endettement.

La réduction du déficit structurel prévue par le Gouvernement, qui s'écartait déjà très significativement des règles européennes, est ainsi revue à la baisse sur la période 2019-2021. Ce choix aura pour conséquence directe de nourrir la divergence de notre trajectoire d'endettement par rapport au reste de la zone euro.

Un second facteur de fragilité tient au manque de documentation de la trajectoire budgétaire, qui ne permet pas réellement au Parlement de porter un jugement sur la crédibilité des engagements pris.

grossière à ce stade, certes, les enjeux budgétaires pourraient donc aller jusqu'à 0,4 point de PIB, en l'absence de mesures de compensation. Peut-être allez-vous nous indiquer, monsieur le ministre, quelles économies réelles permettront de financer ces mesures nouvelles

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui du projet de programme de stabilité pour les années 2019 à 2022, avant sa transmission à la Commission européenne, qui doit intervenir au plus tard demain. Notre commission a souhaité ce débat en séance car il s'agit de la programmation de l'ensemble de nos finances publiques, qui engage la crédibilité de notre pays à l'égard de nos partenaires européens, à quelques semaines du renouvellement des institutions communautaires. Le Parlement ne peut pas en être tenu à l'écart. Ce débat nous laissera cependant sur notre faim. En effet, je cite, « le programme de stabilité a été établi indépendamment des conclusions qui pourront être tirées du grand débat national et constitue le point de référence technique » préalable aux décisions qui seront prises en matière de fiscalité ou de dépense publique. Il est pour le moins singulier que le Gouvernement soumette au Parlement et à la Commission européenne une présentation technique déconnectée des décisions politiques. Mais il est vrai que les ministres étaient dans l'attente des arbitrages présidentiels. Or les arbitrages du Président de la République ont finalement été annoncés jeudi dernier, lors d'une conférence de presse. Outre l'engagement général de ne pas augmenter l'impôt et de réduire « significativement l'impôt sur le revenu, sont annoncées la suppression de niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique, sans autres précisions. Les arbitrages difficiles sur la fiscalité énergétique sont renvoyés à plus tard. Une convention citoyenne serait mise en place en juin. Depuis l'intervention présidentielle, le Gouvernement a annoncé que 15 millions de foyers seraient concernés par la réduction d'impôt sur le revenu, pour un coût de 5 milliards d'euros, en se gardant bien de préciser les contreparties exigées. S'il dit avoir entendu la demande de nos concitoyens d'une plus grande justice fiscale,

En matière de maîtrise de la dépense publique, le Président de la République indique : « Nous pouvons faire aussi bien en dépensant moins et donc supprimer nombre d'organismes inutiles.

En réalité, ce programme, dit « de stabilité », témoigne de la perspective d'une dégradation de nos finances publiques. Celle-ci est due pour partie à la révision à la baisse des hypothèses de croissance l'an passé, le programme de stabilité tablait sur une croissance de 1,9 % en 2019 et de 1,7 % au-delà. Celle-ci est ramenée à 1,4 % sur toute la période. Ce ralentissement n'est évidemment pas sans lien avec l'évolution de l'économie mondiale

Le solde public, qui devait se redresser jusqu'à redevenir légèrement excédentaire en 2022, serait finalement déficitaire de 1,2 point de PIB à la fin du quinquennat. La dette publique atteindrait 96,8 % du PIB, et non 89,2 %. Le déficit structurel resterait à un niveau élevé sur toute la période, tandis que le taux de prélèvements obligatoires serait de 44 % du PIB en 2022, comme en 2019, avec un rebond en 2020 et 2021, que le Gouvernement explique par le « contrecoup » de la transformation du CICE,

sociétés à 25 %, alors même que le taux de prélèvements obligatoires ne devrait pas continuer de baisser dans la trajectoire qu'il présente- mais sans doute est-elle déjà obsolète -et surtout que le financement de ces mesures reste inconnu. Certes, le Gouvernement annonce que la dépense publique sera réduite de 54 % du PIB en 2019 à 52,3 % du PIB en 2022, mais le Président le Président de la République n'a rien annoncé de concret à ce sujet. Quant au programme national de réforme, il mentionne seulement le projet de loi de transformation de la fonction publique. Il est vrai que sont citées la poursuite de la « transformation » de la politique du logement, avec la modification de la base de calcul des APL, qui vient pourtant d'être repoussée, la réforme de l'audiovisuel public, qui n'est pas encore faite, la réduction du volume des contrats aidés, dont on voit mal qu'elle puisse encore s'accélérer, et « la revalorisation maîtrisée de certaines prestations de l'État, notamment des pensions L'ensemble de ces mesures, qui visent parfois les plus modestes, ne permettent pas de dessiner des perspectives d'avenir. Le Président de la République les a d'ailleurs contredites en annonçant une réindexation des pensions de moins de 2 000 euros en 2020 et la fin de toute sous-indexation en 2021. Si l'on regarde les différentes composantes de la dépense publique, on observe que le déficit de l'État restera élevé sur tout le quinquennat. Seuls les excédents des administrations publiques locales, et plus encore des administrations de sécurité sociale, permettraient aux comptes publics de se redresser légèrement, tout en restant déficitaires. Le Gouvernement s'en remet donc à ses partenaires publics pour redresser la barre,

Il y a seulement un an, la trajectoire des comptes publics pouvait sembler prometteuse. La prévision de croissance était de 2 % pour 2018 et de 1,9 % pour 2019. Le déficit public devait s'établir à 2,3 % du produit intérieur brut pour 2019, les comptes publics devant revenir à l'équilibre, voire connaître un léger excédent en 2022, date à laquelle la dette publique était censée passer sous la barre des 90 % du PIB. Mais un an en politique, comme en matière de prévisions économiques, c'est un siècle ! Aujourd'hui, force est de constater que les choses ont changé depuis nos échanges du mois d'avril dernier. La prévision de croissance est désormais de 1,4

Toutefois, la contribution des comptes sociaux, lesquels intéressent plus particulièrement le rapporteur général de la commission des affaires sociales, reste positive sur l'ensemble de la période. Elle s'accroît même en fin de période par rapport à l'année dernière puisqu'elle n'est plus plafonnée à 0,8 % du PIB. Le solde des administrations de sécurité sociale prises dans leur ensemble, les fameuses ASSO, serait ainsi de 0,5 % du PIB en 2019, de 0,8 % en 2020, avant d'atteindre 1 % du PIB en 2021 et même 1,2 % en 2022. Pour le sous-secteur des ASSO, ces chiffres peuvent donc apparaître de prime abord comme une bonne surprise dans un univers globalement moins « rose » pour les finances publiques. Néanmoins, ils interpellent, du fait notamment de l'imprécision des documents d'analyse dont dispose le Parlement. En effet, le détail de la contribution des différents types d'ASSO n'est, lui, pas connu. Or, s'agissant des prévisions que je connais le mieux, correspondant au périmètre des lois de financement de la sécurité sociale, la situation financière tend, elle, à se dégrader, pour des raisons évidentes : une évolution des recettes moins favorable que ce que nous pensions l'an dernier du fait d'une croissance moins forte qu'escompté, et l'effet des mesures prises dans le cadre de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

Il s'agit là d'une évolution un peu contradictoire avec les prévisions du Gouvernement s'agissant des ASSO. De plus, certains chiffres sur lesquels se fonde la prévision du programme de stabilité peuvent également surprendre. Pour prendre l'exemple le plus frappant, le Gouvernement prévoit que les dépenses des ASSO ne progresseraient que de 1,5 % en 2020, contre environ 2 % ces trois dernières années. Monsieur le ministre, sur quels éléments vous appuyez-vous pour prévoir un tel ralentissement en 2020, alors même que nous savons que les retraites seront, au moins en partie, réindexées

Sur cette base, la nouvelle trajectoire financière du régime général et du FSV est-elle compatible avec la fin de la dette sociale pour 2024, comme cela est prévu ?

! Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le 10 avril dernier, le Gouvernement a présenté, en application des règles fixées par le pacte de stabilité et de croissance, et dans le cadre du semestre européen, le programme de stabilité de la France. Deux ans après le changement de majorité, deux ans après le début du travail du gouvernement d'Édouard Philippe, ce programme de stabilité donne un état des lieux précis de la situation des finances publiques de la France et de la trajectoire budgétaire de notre pays. Alors, dans les faits, où en sommes-nous ? Le déficit public a été réduit d'un point de PIB en seulement deux ans : il se situe désormais à 2,5 % du PIB, soit son niveau le plus bas depuis 2006. Pour la première fois depuis 2007, la dette publique a été stabilisée à 98,4 % du PIB, cela en intégrant la dette de SNCF Réseau, représentant 1,7 point de PIB. la dépense publique a décru, en volume, de 0,4 % et son poids dans le PIB est passé de 55 % à 54,4 %, hors crédits d'impôts. Une telle tendance est inédite depuis des décennies. Enfin, les prélèvements obligatoires ont connu une réduction sans précédent.

et la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés représenteront les 16 milliards d'euros supplémentaires. Je crois qu'il faut se satisfaire collectivement de ces chiffres. Il faut s'en satisfaire, en se remémorant les événements politiques et juridiques des deux dernières années.

À ceux-là s'ajoutent 5 milliards d'euros pour rendre sincères les sous-budgétisations de la majorité précédente, sous-budgétisations régulièrement critiquées par la Cour des comptes. Ces chiffres montrent néanmoins l'effort qu'il reste à fournir pour le redressement de la trajectoire des finances publiques de notre pays. Cela a été dit, la réduction du ratio de dépenses publiques

aussi être lus au regard de l'actualité. Cette actualité nous a rattrapés avec force. Elle nous a rattrapés à l'automne dernier, quand les Français ont exprimé une juste indignation et leur impatience face aux problèmes qui les touchent et auxquels nous avions tous collectivement échoué à répondre. Ils ont demandé une baisse plus rapide de la pression fiscale. Eh oui Outre les 32 milliards d'euros de baisses d'impôts déjà engagés, le Président de la République a, lors de sa conférence de presse de jeudi dernier, annoncé une baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes. Elle sera votée en loi de finances pour 2020 et effective dès janvier 2020. Vous avez, monsieur le ministre, précisé les contours de cette baisse. Elle concernera environ 15 millions de foyers, principalement sur la première tranche de l'impôt sur le revenu. Les Français ont aussi demandé plus de services publics, notamment de proximité. Le Président de la République a fait des annonces fortes, avec la création d'un point regroupant l'ensemble des services publics dans chaque canton- il y en a 4 000 en France. Il a aussi annoncé le gel des fermetures d'écoles et d'hôpitaux, qui ne pourront avoir lieu sans l'accord des maires. Avec ces annonces, le Président de la République a fait le choix de répondre à cette colère sourde, ce sentiment de déclassement et d'abandon de nos territoires. Il a aussi, et sans ambiguïté, revu l'objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires.

Nous le dirons très clairement, donner plus de services publics de proximité, c'est une priorité. Limiter à 24 élèves les classes jusqu'au CE1, c'est une priorité dans la lutte contre les inégalités de vie minant notre pays. C'est aussi une urgence pour que notre système éducatif soit à la hauteur. Nous serons clairs également sur ce fait : la baisse de la pression fiscale et le renforcement des services publics devront être financés, tout en respectant notre trajectoire de finances publiques. Nous aurons enfin le débat sur les niches fiscales bénéficiant aux entreprises. Lesquelles ? Il faudra supprimer celles qui n'atteignent pas les objectifs fixés, ... Lesquelles ? ... celles dont l'avantage coût-bénéfice n'est pas favorable, notamment sur les créations d'emplois. Notre pays a besoin d'incitations fiscales à la prise de risque. Il ne faudra toutefois pas céder à la facilité. Réduire les allégements de charges au-delà de 1,6 SMIC ne conduirait-il pas à construire des trappes à bas salaire ? Enfin, le Président de la République souhaite que nous aboutissions, pour le premier trimestre 2020, sur un nouvel acte de décentralisation. Aujourd'hui, toutes les politiques- logement, transport, éducation, sport -sont exercées par plusieurs échelons. C'est incompréhensible Clarifier les compétences, supprimer- enfin ! -les doublons, faire correspondre l'élection à une compétence pour que chacun soit responsabilisé, faire correspondre les services publics aux réalités des territoires : ce chemin sera long, mais il est nécessaire. En conclusion, mes chers collègues, le programme de stabilité dont nous

En tout état de cause, deux ans après l'élection d'une nouvelle majorité, ce programme de stabilité confirme l'efficacité des choix pris par le Gouvernement dont vous faites partie, monsieur le ministre : baisse des prélèvements obligatoires, sortie de la procédure de déficit public et, en même temps, investissements massifs sur la formation des plus éloignés de l'emploi, sur l'école et l'enseignement supérieur. Ces orientations sont confirmées par les annonces récentes du Président de la République. Mais, dans un pays où le ratio des dépenses publiques sur le PIB ne peut dériver, ces mesures devront s'accompagner de réformes profondes de l'appareil de l'État et de l'action publique. Depuis le temps qu'on vous le dit ! Notre groupe sera vigilant à ces choix, dans le respect des préoccupations exprimées par les Français dans le cadre du grand débat.

européen. Comme beaucoup d'entre vous- la plupart, voire tous -, nous sommes profondément attachés au rôle des parlements nationaux. Le contrôle budgétaire et des finances publiques doit être du ressort des représentants élus du peuple, non de technocrates ou des marchés financiers. Ce n'est pas à la Commission européenne de délivrer, ou non, un satisfecit à la politique budgétaire du Gouvernement ; c'est au contraire aux représentants de la Nation d'en définir les choix.

Preuve en est, la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen refusa, en novembre dernier, de transférer ce traité en droit européen, pour cause de non-conformité. En cette période de campagne pour les élections européennes, je veux ici réaffirmer que ce modèle de construction européenne, contraignant les finances publiques, ne répond pas aux attentes légitimes de millions de nos concitoyens européens. Cette construction européenne est, à l'heure actuelle, un échec économique. Plutôt que de contraindre les plans de relance nationaux, le soutien au développement économique, nous agissons pour un développement solidaire et partagé à l'échelle du continent, adossé, notamment, à un nouveau rôle de la Banque centrale européenne. Bien qu'illégitime à nos yeux, la procédure dans laquelle se place le programme de stabilité n'en est pas moins fort instructive. Monsieur le ministre, le débat que nous ouvrons aujourd'hui se place dans un contexte très particulier à plus d'un titre.

Ces situations devraient nous faire réfléchir, vous faire réfléchir. Elles devraient influer concrètement sur la politique économique menée. Face à une croissance atone, pour répondre aux besoins de protection et de service public exprimés par nos concitoyens, par nos concitoyens, la dépense publique et la justice fiscale sont nécessaires, l'une n'allant pas sans l'autre. Néanmoins, le programme de stabilité que vous nous présentez ne tire aucune leçon de la situation, ni du mouvement social en cours ni du ralentissement économique généralisé au sein de la zone euro. Le programme que vous nous présentez est le reflet d'un paradigme, d'un cercle vicieux : baisser les impôts des plus riches et les cotisations des entreprises, d'une part ; baisser les dépenses, d'autre C'est ainsi que vous tentez d'atteindre l'équilibre. Cela, au moins, vous l'affirmez clairement : « la poursuite des efforts en dépense permettrait de financer la poursuite de la baisse des prélèvements obligatoires Ce choix n'est pourtant pas sans conséquences. Nous voulons, ici, alerter l'ensemble des parlementaires et, à travers eux, l'ensemble de nos concitoyens. Ce choix idéologique est injuste socialement et inefficace économiquement. Au regard des données de ce programme de stabilité, il aura, au moins, trois conséquences- particulièrement injustes -que je tiens à souligner. Premier point, sur la durée, le cap fixé est de faire baisser la dépense publique de 3 points à l'horizon de 2022. Un tel objectif ne sera pas neutre pour les politiques publiques. Comme la Cour des comptes le soulignait dans un rapport de juin 2017, il conduira à réaliser près de 80 milliards d'euros d'économie. En somme, c'est véritablement un nouveau plan d'austérité que vous proposez aux Français. Deuxième point, la poursuite des exonérations de cotisations sociales met en péril l'équilibre de la sécurité sociale et son financement par les revenus du travail. Elle conduit à une fiscalisation toujours plus importante de notre système de protection sociale. La montée en charge de la CSG fera reposer sur tous les citoyens ce qui devrait dépendre des revenus du travail. Elle conduira, lentement, mais sûrement, à faire reculer la gestion par les partenaires sociaux et, donc, la démocratie sociale. point, ce programme de stabilité est porteur de choix en matière de politiques publiques. Il faut le dire à nos compatriotes, il privilégie les coupes dans les services publics, dans la protection sociale, pour favoriser un resserrement étroit sur les missions régaliennes et les opérations militaires extérieures, par exemple. Monsieur le ministre, ce que vous détruisez, c'est l'État social ; ce que vous construisez, c'est l'État gendarme. Ce programme de stabilité marque, par ailleurs, l'échec de la politique économique que vous menez depuis deux ans. Le symptôme immédiat en est le ralentissement de la croissance. Je voudrais me focaliser sur un autre point : la poursuite du CICE et sa transformation en baisse de cotisations sociales sont, à ce titre, tout à fait exemplaires.

et le déficit public : seuls nos créanciers, les marchés financiers, sauront s'en féliciter. Là encore, les cadeaux que vous faites aux grandes entreprises gagent l'avenir de la Nation dans son ensemble. Enfin, dans la lignée de l'avis adopté voilà peu par le Conseil économique, social et environnemental sur votre programme de stabilité et de réforme, je souhaiterais pointer les sujets qui ne sont pas abordés. Ces impasses définissent, tout autant que vos coupes budgétaires, la nature de la politique que vous entendez mener. La transformation de l'action publique que vous préconisez ne mentionne même pas l'intérêt général et procède avant tout d'une logique comptable. Les partenaires sociaux n'ont pas été consultés. La question du logement n'est pas abordée dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Vous comprendrez, monsieur le ministre, que nous sommes extrêmement inquiets à la lecture du programme de stabilité que vous nous présentez. n'est pas à la hauteur des défis de relance et de lutte contre la récession que la France et l'Europe doivent affronter. Il organise un transfert de fiscalité des entreprises vers les contribuables dans leur ensemble. À l'image de la conférence de presse du Président de la République la semaine dernière, il ne répond pas du tout à la profonde crise sociale et politique que notre pays traverse. La parole

L'an dernier, cette question avait fait l'objet d'une déclaration du Gouvernement au sens de l'article 50-1 de la Constitution. C'est toujours un rendez-vous indispensable, surtout à quelques semaines des élections européennes, où nous pouvons prendre du recul sur l'année écoulée et tracer les perspectives du prochain cycle budgétaire. Nous étions sortis de l'audition du président du Haut Conseil des finances publiques, Didier Migaud, avec l'impression parfois embarrassante d'un manque de visibilité inédit sur les prévisions économiques à court et moyen termes. Nous avons pourtant l'habitude des prévisions incertaines en matière économique, que le rapporteur général aime souvent à comparer à la science météorologique. Pourtant, cette année, les différents indicateurs dont nous disposons peinent à tracer une voie, tant sont nombreux les points d'interrogation, à commencer par l'état du commerce international. La chute brutale du commerce mondial à la fin de 2018, après des années de stabilisation et de remontée depuis la crise de 2008, est le phénomène le plus spectaculaire de ces derniers mois plus que les incertitudes liées au Brexit, la situation de l'Italie ou encore la crise des « gilets jaunes » chez nous, même si je ne sous-estime bien évidemment pas ces autres sujets. Dans ce contexte, l'économie française bénéficie, pour ainsi dire, de la force de ses faiblesses. Importatrice nette depuis plusieurs années, donc moins exposée que ses voisines allemande, italienne ou néerlandaise, elle est logiquement moins affectée par un ralentissement soudain des échanges mondiaux. Mais cet avantage, relatif et conjoncturel, ne doit pas faire oublier les difficultés structurelles en termes d'offre, de production, de compétitivité, auxquelles le Gouvernement s'efforce depuis bientôt deux ans de répondre. De plus, nous restons vulnérables à une hausse des prix des carburants, qui a été, ne l'oublions pas, l'un des facteurs déclencheurs du mouvement des « gilets jaunes désormais plus contraint, il faut donner crédit au Gouvernement d'avoir cherché à améliorer la maîtrise des comptes publics, avec un déficit ramené sous la barre des 3 % du PIB en 2017 et 2018, et une certaine stabilisation de l'endettement public un peu au-dessous de 100 % du PIB, un niveau certes élevé. Le véritable risque pourrait venir de l'endettement privé. Alors que l'endettement des ménages a été à l'origine de la crise financière de 2007-2008 aux États-Unis et dans certains pays européens, l'endettement privé, des entreprises et des ménages, est aujourd'hui plus élevé en France que la totalité de la dette publique. Il est vrai que la politique de taux bas, voire nuls, de la Banque centrale européenne depuis plusieurs années facilite beaucoup l'accès au crédit et que, associée à une inflation faible, elle encourage les agents privés à s'endetter. Les niveaux désormais atteints devraient conduire à une certaine vigilance, en particulier en ce qui concerne les entreprises. D'après le journal, en 2015, la dette des entreprises équivalait à 125 % du PIB, soit 30 % de plus que la dette publique. Si la dette peut être un levier pour investir et faire croître l'économie, les crises passées nous ont appris qu'elle comporte des risques contre lesquels il est essentiel de se prémunir. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer quel suivi votre administration effectue de ce phénomène et quel est le niveau de coordination avec les autorités monétaires européennes ? Pour ce qui concerne la stratégie de gestion des finances publiques, l'année 2019 devait de toute façon être marquée par la transformation du CICE en réduction de cotisations sociales. À cela s'ajoutent les mesures d'urgence votées à la veille de Noël dans le contexte que nous connaissons. Je note que le Gouvernement a d'ores et déjà décidé de recettes supplémentaires dans le projet de loi sur la taxation des services numériques que nous examinerons prochainement. Son article 2 déroge à la trajectoire de réduction de l'impôt sur les sociétés à l'horizon de 2022, pour un rendement estimé à quelque 1,7 milliard d'euros. Je n'oublie pas non plus, évidemment, l'impact à venir des dernières annonces du Président de la République, dont nous attendons maintenant de connaître précisément les contours législatifs. Toutes choses étant égales par ailleurs, le solde public devrait s'améliorer automatiquement en 2020 du fait de la disparition de la mesure ponctuelle liée au CICE. Mais alors, c'est l'environnement international qui reste assez incertain. Il me semble qu'une des conclusions essentielles à tirer du mouvement des « gilets jaunes » et du grand débat national est une exigence, à la fois, de justice fiscale et de meilleur usage des deniers publics. Beaucoup de Français refusent davantage d'impôts, cela paraît clair. Mais ils ne veulent pas nécessairement moins de services publics. En revanche, ils souhaitent que chaque euro dépensé par la puissance publique, qu'il s'agisse

sont en adéquation avec les données du moment. Elles sont réalistes et claires. Le groupe Union Centriste tient à le saluer. Mais, nous le savons, les aléas sont nombreux- sur le plan mondial, européen et national. Qui pourrait aujourd'hui prédire la stratégie commerciale américaine à l'approche des élections de 2020 et les conséquences de ses à-coups douaniers et tarifaires sur l'économie européenne et française ? ? de l'issue du Brexit et de la nouvelle configuration de la politique européenne, au sortir des élections du 26 mai ? Comment mesurer avec précision l'impact des orientations fixées par le Président de la République à l'issue du grand débat ? la suppression de la taxe d'habitation, d'un coût supérieur à 10 milliards d'euros, est-elle intégrée à la trajectoire des finances publiques que vous nous présentez ? Il faut l'espérer ! Pensez-vous, monsieur le ministre, que ces aléas pourraient vous amener à réviser le programme de stabilité ? Quoi qu'il en soit, malgré ces incertitudes, notre pays doit garder le cap : le cap de la bataille de l'emploi, dont les premiers résultats sont encourageants ; le cap de la nécessaire transformation de notre pays et de son adaptation aux enjeux du XXI siècle le cap du redressement des comptes publics, qui doit rester une priorité. Cet objectif exige de chacun d'entre nous un devoir de cohérence et de responsabilité. On ne peut pas réclamer simultanément la baisse des impôts, la réduction du déficit, la diminution de la dette, sans préciser avec quels moyens nous organiserons la présence des services dans les territoires, alors même que nous devons faire face à l'allongement de la durée de vie et au phénomène de dépendance qui l'accompagne. Pour ma part, je considère que la baisse des prélèvements obligatoires ne doit pas être un objectif aveugle. Oui à la baisse de l'impôt sur le revenu pour les premières tranches et les classes moyennes ! Oui à la baisse de l'impôt sur les sociétés pour gagner le pari de l'innovation, de la recherche, de l'investissement, de l'emploi aussi, à une juste taxation des GAFA ! À cet égard, nous soutenons votre position en faveur de la création d'un impôt minimum mondial ! Et oui à une lutte efficace, plus efficace, contre l'évasion fiscale et à l'encadrement de l'optimisation fiscale : nous pouvons faire mieux Pour susciter l'adhésion de nos concitoyens- mieux, pour qu'ils soient partie prenante d'une dynamique collective -, la mise en oeuvre des réformes doit avoir, pour principale boussole, la recherche d'une plus grande équité. Monsieur le ministre, la nécessaire transformation de notre société et le redressement des comptes publics doivent s'appuyer sur une exigence permanente de justice sociale, de justice fiscale, de justice territoriale.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chaque année, le programme de stabilité fera l'objet d'une attention toute particulière de la part de la Commission européenne, ainsi que des autres pays européens. Et pour cause : du fait du poids économique de la France, la trajectoire de nos finances publiques revêt une importance singulière aux yeux de nos partenaires. Comme chaque année, le programme de stabilité français suscitera chez eux de nouveaux espoirs. Mais les gouvernements précédents ont pris la mauvaise habitude de décevoir ces espoirs, si bien que la crédibilité de la France s'en est trouvée écornée. Durant de trop nombreuses années, nous avons inlassablement rejoué la même farce : au printemps, nous nous targuons de notre rigueur future et, à l'automne, nous nous accommodons de notre désinvolture. Cette année encore, ce document fera donc éclore les mêmes espoirs printaniers. Cependant, nous aurions tort de ne pas apprécier ce programme de stabilité à sa juste valeur. Il faut le dire, la trajectoire qu'il présente nous remet sur de bons rails. C'est comme si nous entrions dans une gare : l'horaire du train nous convient ; encore faut-il qu'il arrive à l'heure Les principaux indicateurs devraient ainsi repasser à l'orange : réduction du déficit à 2,3 % du PIB en 2019, abstraction faite de la bascule comptable du CICE, soit la troisième année consécutive sous la barre des 3 maîtrise de la dépense publique à 0,2 % par an, soit l'équivalent de 3 points de PIB sur l'ensemble du quinquennat ; baisse de 1,4 point de PIB pour les prélèvements obligatoires sur la même période ; inversion de la courbe de la dette, avec, pour la première fois depuis des décennies, une diminution de son volume global De même, les prévisions actualisées de croissance, bien qu'elles aient été revues à la baisse, confirment une tendance solide, aux alentours de 1,4 % pour 2019 et 2020, au-dessus de la moyenne de la zone euro, portée notamment par une consommation vigoureuse. Pour réaligner durablement la trajectoire de nos finances publiques sur les objectifs du pacte de stabilité, il faut nécessairement revenir aux fondamentaux. Les réformes annoncées peuvent aller dans le bon sens, mais les efforts portés à la fin du quinquennat nous interrogent. De plus, tout ne dépend pas de nous et nombreux sont les nuages qui assombrissent ces perspectives de croissance : incertitudes liées au Brexit et à la possibilité d'un ; tensions commerciales avec les deux géants mondiaux ; tentations protectionnistes chez certains de nos partenaires, notamment européens. Hélas, mes chers collègues, rien de nouveau sous le soleil, et les mauvais augures d'une dégradation généralisée du commerce international vont bon train. Mais en économie, c'est bien connu, quand la confiance disparaît, la crise survient Tâchons donc de reprendre confiance en nous-mêmes pour inspirer confiance aux autres. Nous ferons ainsi entendre les revendications françaises au niveau européen, par exemple sur les questions climatiques dans le cadre des négociations à venir pour un accord commercial avec les États-Unis. Mes chers collègues, ce programme de stabilité n'est ni une cure d'austérité ni une sinécure : il nous permet simplement de respecter les engagements que nous avons pris au niveau européen. Pour nous préparer à une prochaine crise, rien ne sert de prédire un éventuel relèvement des taux ou une hypothétique crise de la dette : il faut continuer d'assainir nos comptes publics, afin de nous prémunir de temps moins cléments. Pourtant, nous aurions vraiment tort de croire que le danger ne peut venir que de l'extérieur. La crise des « gilets jaunes » nous rappelle qu'un équilibre est toujours fragile et que la stabilité ne se laisse pas facilement programmer. Le Gouvernement l'a réaffirmé à l'issue du grand débat : parce que l'exaspération fiscale est à son comble, il faudra baisser les prélèvements obligatoires et, pour baisser les prélèvements obligatoires, il faudra encore réduire les dépenses publiques. Aussi, les annonces faites par le Président de la République, notamment concernant la baisse de l'impôt sur le revenu, devront-elles s'inscrire dans le strict respect de cette trajectoire. Il nous faudra persévérer pour restaurer la crédibilité des programmes de stabilité français. Il y va, à Paris comme à Bruxelles, de la crédibilité des responsables politiques politiques français. Dans la crise de confiance que nous traversons, nous devons démontrer que nous pouvons tenir nos engagements. Les difficultés sont trop nombreuses, à l'intérieur comme à l'extérieur de nos frontières. Mais c'est le chemin qui doit nous ramener dans les clous de Maastricht, avec, en ligne de mire, une dette ramenée sous la barre des 60 % du PIB. Sans aller jusqu'à l'austérité, nous aurons besoin de rigueur. Comme l'a dit Paul Valéry, « la plus grande liberté naît de la plus grande rigueur Mes chers collègues, attachons-nous à tenir rigoureusement un programme de stabilité. C'est notre devoir à l'égard des générations futures. Mais c'est aussi la première étape d'une réflexion de fond, qui doit nous amener à repenser la place et le rôle de l'État dans la société. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, avant tout, je tiens à remercier le président de notre commission des finances et notre rapporteur général d'avoir pris l'initiative d'organiser ce débat au Sénat, puisque le Gouvernement ne l'avait pas jugé utile ... Certes, ce débat est percuté de plein fouet par l'actualité, mais c'est ainsi.

Mais ce n'est pas tout : il y a à la fois les mesures annoncées et les déclarations du Président de la République, qui laissent perplexe. Lors de sa conférence de presse, il a en effet annoncé son intention de ne pas tenir l'objectif de suppression de 50 000 postes dans la fonction publique d'État. Quel est donc le nouvel objectif ? Quelles seront ses conséquences sur la trajectoire des finances publiques ? Nul ne le sait. S'y ajoute une autre réforme majeure pour l'équilibre à venir de nos finances publiques : celle des régimes de retraite. Coincés par la promesse électorale de ne pas toucher à l'âge de départ, vous avez perdu des mois, et certainement la confiance des partenaires sociaux, en laissant finalement entrevoir votre point d'arrivée un départ toujours possible à 62 ans, mais avec une décote. Ce sera d'ailleurs, manifestement, votre argument majeur : la liberté de choisir entre obtenir une pension avec décote ou travailler plus longtemps. Quel manque de courage de courage ! Surtout, comment anticiper les effets d'un tel système sur l'équilibre du futur régime, puisqu'il dépendra de ce choix laissé aux Français ? Seule une décote importante les contraindra à travailler plus longtemps. Sur quelles hypothèses sera donc bâtie la réforme ? Quel sera son impact sur nos finances publiques ? Nous ne le savons toujours pas. Je pourrais également parler de nos collectivités territoriales, qui depuis 2014 ont été largement mises à contribution au titre du redressement des finances publiques et qui sont- rappelons-le ici, au Sénat -les bons élèves de la classe. elles sont de nouveau sollicitées par le Président de la République depuis jeudi dernier, pour l'ouverture de maisons de services publics dans tous les cantons de France et la réduction du nombre d'élèves par classe.

: si l'État ne réduira pas de 50 000 le nombre de ses fonctionnaires, les collectivités territoriales sont priées de bien vouloir tenir l'objectif de 70 000 postes en moins. Comment feront-elles pour concilier tout cela ? Avec quelles ressources, puisque vous avez repoussé à l'automne la réforme de la fiscalité locale ? Elles ne le savent toujours pas.

? Au-delà des chiffres, le plus important est certainement l'abandon pur et simple de l'objectif de retour à l'équilibre de nos comptes publics en 2022. Il en va donc de ce quinquennat comme de celui de François Hollande, toutes proportions gardées ... Moins de deux ans après son commencement, on change de politique et l'on repousse encore et toujours le retour à l'équilibre des finances publiques. En 2012, François Hollande le promettait pour 2015 : on connaît la suite. En 2017, vous le promettiez pour 2022 : c'est terminé. Le point commun de ces deux tournants, c'est bien sûr le ras-le-bol fiscal. Certes, monsieur le ministre, vous n'avez pas assommé les Français de 30 milliards d'euros d'impôts nouveaux, comme le fit le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, cher Claude Raynal, ...

Sur ce point, vos prévisions à la baisse semblent prudentes, mais le sont-elles assez ? Comme ce fut le cas en 2008 et 2009, la situation en Allemagne se dégrade plus vite qu'en France. Certains s'en réjouissent. Mais souvenons-nous, mes chers collègues, que cette situation est d'abord due au fait que l'Allemagne exporte beaucoup et que nos exportations sont bien moindres, ce qui est l'une l'une de nos faiblesses. Monsieur le ministre, vous anticipez effectivement ce ralentissement, mais n'êtes-vous pas encore trop optimiste ? Si, dans ce contexte, les mesures de décembre et celles de jeudi dernier soutiendront opportunément la consommation et le pouvoir d'achat des ménages, elles constituent certainement- il faut en avoir conscience -la dernière cartouche de votre gouvernement, sauf à laisser s'emballer le déficit et la dette, en cas de coup dur, bien au-delà des 100 % du PIB. ans après la crise de 2008, alors que la plupart de nos partenaires européens ont rétabli ou grandement amélioré le solde de leurs comptes publics, la France est toujours à la traîne, au moment même où les nuages s'amoncellent de nouveau. La petite phrase du Président de la République- » l'important ce n'est pas la comptabilité, mais la transformation de l'État » -est un renoncement inquiétant, qui s'apparente à un « après nous, le déluge », d'autant que, pour la transformation de l'État, nous attendons toujours de voir. Encore une fois, il aura été démontré que les erreurs commises en début de quinquennat ne se rattrapent pas et se paient cash. Il ne nous reste plus qu'à prier le ciel, pour que le trou d'air de la croissance ne soit pas trop violent ; que le prix du pétrole ne remonte pas trop ; pour que la guerre commerciale ouverte par les États-Unis trouve enfin un terme ; pour que le Brexit se dénoue sans trop de dommages ; et pour que les taux d'intérêt restent relativement bas. Que d'incertitudes Que d'incertitudes ! Plus le temps passe, plus le sort de la France dépend fortement d'éléments extérieurs, plutôt que de ses propres choix. Voilà où nous en sommes, deux ans à peine après l'avènement du « nouveau monde

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues,

Pourtant, les travaux conduits par notre commission des finances laissent à penser qu'un « hardBrexit » pourrait se traduire par une perte de 1 point de PIB pour la France, et qu'un Brexit négocié aurait également des conséquences, tout comme un report du Brexit.

Si le Haut Conseil des finances publiques a pu qualifier le scénario macroéconomique de ce programme de stabilité de crédible, je reste très réservé, pour les raisons indiquées. Du fait de cette conjoncture très particulière, il eût très certainement été opportun de solliciter la Commission européenne pour obtenir d'elle un report de quelques jours pour la remise du document, afin de prendre en compte ces éléments. Après l'épisode du projet de loi « gilets jaunes », débattu dans des conditions pour le moins baroques, le Gouvernement réitère et transmet au Parlement un document de toute évidence très approximatif. Nous en prenons acte. J'en viens maintenant au fond. En tant que tels, les éléments mis en avant dans le programme de stabilité ne sont pas à proprement parler originaux, mais ils méritent à certains égards d'être évoqués, car la présentation qui en est faite me semble lacunaire. La prévision de croissance pour 2019 et les années suivantes s'établit à 1,4 % du PIB, soutenue principalement par la consommation des ménages, traditionnellement plus favorable à la France qu'à ses principaux partenaires.

également sur une amélioration notable de la balance commerciale de la France. Néanmoins, il convient de rappeler, d'une part, que la France reste largement déficitaire en la matière, et, d'autre part, que la remontée en cours des prix du baril par rapport aux prévisions établies dans le document, tout comme l'importance accrue de la consommation des ménages, risque de conduire à une dégradation de cette balance commerciale. Monsieur le ministre, je ne peux que vous inviter à la plus grande prudence sur ce point ; je ne doute pas que vous en fassiez comme le document l'établit, la demande mondiale adressée à la France devrait perdre 1 point en 2019, pour s'établir à 2,7 %. Cette décélération, plus marquée que celle du commerce mondial, témoigne des risques pesant sur le solde commercial du pays. Les prévisions d'amélioration de ce solde à partir de 2019 et 2020 m'apparaissent, en ce sens, très hypothétiques. En matière de croissance, il convient également de noter les aléas frappant le programme de stabilité, liés aux difficultés tant européennes- Brexit, montée de l'euroscepticisme et du populisme

Je ne peux que me satisfaire de mesures qui accroissent le pouvoir d'achat et reviennent pour partie sur vos politiques profondément inégalitaires. Ainsi, il est amusant de lire : « La consommation des ménages serait fortement soutenue en 2019 par les mesures de soutien au pouvoir d'achat, notamment celles décidées en décembre. Pour un peu, on croirait à une volonté politique, et non à ce qui fut une retraite en désordre face au mécontentement de la rue ! Toutefois, à ce stade du moins, cette action est menée au détriment des finances publiques, dans la mesure où les dispositions annoncées ne sont, à ce jour, que très imparfaitement financées. Ce n'est pas la taxe sur les services numériques, qui sera soumise à notre examen le mois prochain, qui permettra de trouver 11 milliards d'euros par an, auxquels s'ajoutent les montants liés aux dernières décisions, pour un total proche de 20 milliards

ont des conséquences : refuser d'assumer cette mesure et de l'inclure dans vos calculs ne la rend pas moins coûteuse pour les finances publiques. De plus, même si elle est ponctuelle, elle fait de la France le seul pays européen à se situer cette année au-delà des 3 % de déficit public. Encore bravo !

de progression en volume des dépenses publiques sur toute la durée du quinquennat. Certes, en 2018, une inflation particulièrement élevée a permis d'y arriver. l'échelle du quinquennat, l'ambition est passée de 0 % en volume en moyenne à 0,2 %, toujours en moyenne, et que nous commençons par 0,4 % cette année, ce qui augure mal de votre capacité à tenir cet engagement. De plus, je rappelle une nouvelle fois que le gouvernement Philippe n'a rien engagé de neuf depuis deux ans. Il se contente de poursuivre une démarche vertueuse amorcée durant le quinquennat précédent,

Sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres, vous faites donc largement moins bien que vos prédécesseurs. Au contraire, loin d'être plus vertueuses que celles des gouvernements précédents, vos politiques ont accru les inégalités. Les allégements d'impôts et de taxations décidés pour le premier décile de la population, voire pour le premier centile, accroissent les disparités et contreviennent à votre objectif de rééquilibrage des comptes publics, sans que les études disponibles montrent un véritable différentiel en matière d'investissement, qui serait

J'attends d'ailleurs avec impatience l'aboutissement des travaux du Sénat en la matière. Je ne doute pas que vous aurez alors la lucidité de réorienter votre politique. La seule certitude dont on dispose, c'est que les très riches ont été les grands gagnants de votre politique fiscale. Quant aux prévisions à plus long terme, il me semble risqué, du fait des grandes incertitudes macroéconomiques et politiques de la période, de donner trop de crédit à des prévisions n'intégrant que de manière marginale ces risques. J'observe cependant que, comme souvent, les deux dernières années du programme sont celles des plus gros efforts ... Prière d'y croire ! Ah, ça ... Pour nous éclairer, rappelons que, l'année dernière, le programme de stabilité prévoyait un solde public nominal de-0,9 % en 2020. Cette année, vous nous parlez de-1,2 % en 2022. Enfin, le document évoque la problématique de la gouvernance budgétaire et la juge « pleinement opérationnelle pleinement opérationnelle ». Or le Parlement travaille bien souvent sur la base d'hypothèses mal assurées, voire de mesures non évaluées, et les éléments statistiques utiles ne sont pas toujours transmis aux parlementaires, par exemple en matière d'évaluation des dépenses fiscales.

Dans sa construction, il part du postulat que la France souffre de faiblesses structurelles en matière d'emploi, de travail et d'insertion, ce malgré un taux de prélèvements obligatoires très élevé et un modèle social coûteux, qui permet de contenir les inégalités, mais pas de les corriger. Je tiens à le dire clairement : toutes les analyses macroéconomiques publiées permettent d'affirmer que les inégalités dans notre pays, si elles tendaient à se résorber durant le quinquennat précédent, progressent de nouveau, du fait notamment des allégements de la fiscalité pesant sur les plus fortunés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai retenu de mes années étudiantes que tenir compte des remarques du correcteur permettait de progresser pour le devoir suivant. Assez naturellement, j'ai donc relu l'évaluation du 25 mai 2018 du Conseil européen portant sur le programme national de réforme de la France pour 2018 et sur le programme de stabilité de la France pour 2018. Très bien ! Ledit Conseil formule trois recommandations à l'élève France pour améliorer ses performances macroéconomiques. La première a particulièrement retenu mon attention : « Veiller à ce que le taux de croissance nominale des dépenses publiques primaires nettes ne dépasse pas 1,4 % en 2019, ... Raté ! ... ce qui correspondrait à un ajustement structurel annuel de 0,6 % du PIB » utiliser les recettes exceptionnelles pour accélérer la réduction du ratio d'endettement public » ; « réduire les dépenses en 2018 et pleinement préciser les objectifs et les nouvelles mesures nécessaires dans le contexte de l'Action publique 2022, afin qu'ils se traduisent en mesures concrètes de réduction des dépenses et de gain d'efficience dans le budget 2019 » ; et « uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite pour renforcer l'équité et la soutenabilité de ces régimes vous ne serez pas étonné que, en tant que représentant du Sénat au sein du comité Action publique 2022, je me sois particulièrement intéressée à la déclinaison opérationnelle du chantier de transformation de l'action publique. Vous devez également savoir à quel point j'ai été déçue par le résultat et la conduite de ces travaux, alors même que je m'étais engagée avec enthousiasme dans la démarche. Je note que les termes « Action publique 2022 » ne figurent nulle part dans le programme de stabilité de la France pour 2019, leur accordait dix mentions, ainsi qu'un encadré aux pages 48 et 49. Dans le programme national de réforme 2018, Action publique 2022 était la source des réponses au deuxième axe du quatrième défi, « transformer l'État et restaurer l'équilibre de nos finances publiques Dans la version 2019 de ce programme, si l'on en croit le tableau de la page 124, l'action de transformation est en marche : « transformation des administrations centrales, déconcentration, refonte du cadre de gestion publique, nouveau contrat social, mise en place d'un suivi de l'exécution à haut niveau, révision de la gestion du parc immobilier de l'État, nouveaux services publics de proximité sur le territoire » ... soit « 75 % des recommandations du comité Action publique 2022 », du moins, vous me permettrez de le préciser, après intervention de la direction interministérielle de la transformation publique dans l'écriture du rapport final. À cette même page 124, on peut lire : « Les transformations issues d'AP 2022 vont notamment se traduire par des baisses du nombre d'emplois publics, déjà mises en oeuvre par les lois de finances pour 2018 et 2019. » Cette affirmation ne manquera certainement pas d'étonner les analystes de la Commission européenne, car elle apparaît en décalage avec la réalité, comme l'a révélé, données chiffrées à l'appui, l'iFRAP. En effet, la baisse annoncée de 4 164 postes en équivalents temps plein coïncide avec une augmentation du plafond d'emplois cumulé de l'État et de ses opérateurs de 1 322 postes entre 2018 et 2019.

promesse de campagne ! -, s'il n'était pas tenable au regard de la sortie du grand débat. Les effets annoncés du programme Action publique 2022 ne sont pas là : entre les versions 2018 et 2019 du programme de stabilité, la baisse des dépenses publiques est moindre de 42 milliards d'euros. En douze mois, l'excédent de 0,3 point de PIB, soit 7,9 milliards d'euros, en 2022 a laissé place à un déficit de 1,2 point. Avant même les dernières annonces du Président de la République, la baisse de la dépense s'est donc dégradée de 1,5 point de PIB.

Ces générations, ce sont celles de mes enfants et de mes petits-enfants. Je m'en sens donc responsable. Au cours des vingt dernières années, dans seize pays de l'Union européenne, la diminution des dépenses publiques a été supérieure à 3 points de PIB potentiel sur cinq ans. Un tel effort est donc réalisable. C'est la voie dans laquelle nous devons nous engager pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, pour une croissance économique « intelligente, durable et inclusive ». À cette fin, des choix courageux s'imposent : il s'agit, par exemple, de dire aux Français qu'ils devront travailler plus longtemps

de venir débattre avec vous dans le cadre de la semaine de contrôle du Parlement pour vous présenter le programme de stabilité pour 2019-2022, même si cette présentation m'a obligé à quitter le séminaire gouvernemental. Après tout, en quittant un séminaire pour une thébaïde, je ne perds pas au change ! Je vous présente ce programme dans un contexte économique international préoccupant, par le ralentissement de la croissance mondiale, souligné par tous mes interlocuteurs lors des réunions de printemps du FMI à Washington, du président de la Réserve fédérale américaine jusqu'à la présidente du FMI en passant par le président de la Banque centrale européenne. Deux facteurs de risques doivent notamment appeler notre vigilance. Le premier est constitué par les risques de nature politique, dont nous sommes entièrement responsables, avec l'augmentation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais également entre les États-Unis et l'Europe. J'ai eu l'occasion de dire à mes interlocuteurs américains, qui n'avaient que ce mot à la bouche,

C'est ce qui m'a amené à prendre des décisions de précaution dans le cadre du Haut Conseil de stabilité financière. Ces risques de tensions commerciales, cet endettement excessif, ajoutés aux incertitudes politiques liées au Brexit, créent un environnement économique international moins favorable qu'il y a quelques mois. C'est ce contexte, avec le ralentissement marqué dans la zone euro, en particulier en Allemagne et en Italie- qui est en récession, qui m'a conduit à proposer un nouveau contrat de croissance à mes partenaires de la zone euro et je recommencerai dans quelques jours. Ce partenariat et ce contrat de croissance

une réforme ambitieuse de l'indemnisation du chômage d'ici à quelques semaines, indispensable pour introduire plus de justice et plus d'efficacité dans le retour à l'emploi ; une réforme des retraites qui changera radicalement le système français, avec un système de retraite par points, et qui permettra d'égaliser les conditions entre le secteur public et le secteur privé, car c'est aussi une question de justice et d'équité profondément attendue par nombre de nos compatriotes une transformation de la fonction publique. Tel est le programme qui est devant nous et qui sera poursuivi avec la même constance et la même détermination. Cela nous autorise à demander aux États qui le peuvent d'investir davantage pour lutter contre le ralentissement de la croissance mondiale et de la zone euro. J'estime que l'Allemagne, les Pays-Bas et d'autres États de la zone euro disposent des marges de manoeuvre nécessaires pour cela. La zone euro, cela ne peut pas être le chacun pour soi, le « vous devez faire des transformations, vous devez faire des réformes, vous devez vous adapter, mais nous, nous ne bougeons pas ». À partir du moment où la France respecte ses engagements de transformation économique,

nous avons eu une réaction responsable, nous avons mis en place de nouveaux instruments, mais ceux-ci ne sont pas suffisants ni pour faire face à une éventuelle crise économique ou financière ni pour accélérer la convergence indispensable entre les économies des États membres de la zone euro. Or une zone monétaire unique dans laquelle nous partageons la même monnaie, mais où les économies divergent, les économies divergent, risque fort de disparaître un jour. Il est donc temps que nous accélérions les décisions nécessaires pour consolider la zone euro et notre monnaie unique afin d'en faire une monnaie de référence sur la scène internationale.

pour laisser notre marché à des investisseurs étrangers, fussent-ils américains, mais d'abord pour le profit de nos entreprises, de nos industries financières ou manufacturières et de nos consommateurs. Il est temps que nous achevions l'union des marchés de capitaux, c'est cela qui nous permettra d'investir, de faire grandir nos entreprises et d'avoir des géants dans les technologies de pointe, comme les Américains ou les Chinois ont su en faire émerger. Il est temps que nous mettions en place un budget de la zone euro pour partager les investissements et pour faire face à une éventuelle crise économique. Je le dis avec beaucoup de gravité : nous ne pouvons plus

donne des résultats et nous devrions tous, ici, nous en féliciter, quelle que soit notre appartenance politique, parce que nous nous portons mieux avec une France qui réussit qu'avec une France qui échoue. S'agissant de nos engagements en matière de déficit public, je veux rassurer Jérôme Bascher : je suis heureux quand nous respectons nos engagements européens et malheureux quand nous ne les respectons pas, parce que je considère que cela affaiblit notre voix sur la scène internationale, alors que celle-ci est absolument décisive. La France

ouvert plus d'entreprises industrielles que nous n'en avons fermé. La réindustrialisation est donc amorcée. Je ne vous dis pas que tout cela est suffisant ou satisfaisant ; je vous dis simplement que nous tenons le bon bout, que nous sommes dans la bonne direction

que nous pourrions nous résigner à laisser la dette française croître et je ne partage pas les analyses de certains économistes qui nous disent : « Ne vous inquiétez pas pour la dette, les taux d'intérêt sont faibles, les conditions de remboursement sont meilleures, vous pouvez donc continuer à vous endetter. » Je considère qu'il est crucial de continuer à nous battre contre la dette ; dès que des marges de manoeuvre se feront jour, je souhaite qu'elles soient consacrées à la réduction de cette dette publique française, qui est aujourd'hui stabilisée.

Ce n'est pas un reproche envers qui que ce soit, et certainement pas envers ceux qui ont un travail, qui sont productifs et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur emploi.

donc impératif que nous créions plus de richesses et que nous accroissions le volume global de travail dans notre pays. La solution passe par le travail ; la meilleure réponse au problème du pouvoir d'achat, au problème de la pauvreté, c'est le travail et l'emploi pour tous les Français : travailler plus, travailler mieux et, surtout, travailler tous. Cela me paraît être la bonne orientation pour notre pays, celle qui a été rappelée avec beaucoup de force par le Président de la République. C'est dans ce contexte que nous présentons le programme de stabilité que vous avez commenté au cours de ce débat. Le déficit sera réduit et maintenu sous les 3 %, c'est un engagement que nous prenons et que nous tenons.

2,3 %, inférieur aux 3 % de la règle européenne. Nous visons un déficit de 2 % en 2020 et de 1,2 % à la fin du quinquennat, en 2022. Sur la dette, je rappelle que, si des marges de manoeuvre supplémentaires apparaissaient, notamment en raison d'une croissance plus forte que prévu, elles devraient être consacrées en priorité au désendettement de l'État.

qui ont été les premiers à payer la facture, au moment même où l'on commençait à l'alléger pour les entreprises. Ce n'est dès lors que justice d'entendre ce cri poussé par beaucoup de nos compatriotes : « Nous voulons vivre dignement de notre travail et, pour cela, nous voulons que les impôts entendu avant vous ! Je dis bien « continuent à baisser », puisque nous avions déjà commencé à baisser les impôts des Français avec la taxe d'habitation, avec la suppression de la cotisation assurance maladie ou assurance chômage. Les impôts vont donc continuer à baisser. L'impôt sur le revenu sera réduit, le Président de la République l'a indiqué, de 5 milliards d'euros et les Français bénéficieront de cette baisse dès le 1 janvier 2020. Je souhaite que ces impôts baissent massivement pour les personnes qui travaillent, en particulier pour les classes moyennes, surtout pour les classes moyennes modestes de la première tranche à 14 %. Plus de 15 millions de foyers fiscaux qui travaillent seront donc concernés. Le Président

comme à la tribune de l'Assemblée nationale : si nous voulons baisser durablement les impôts, il faut aussi baisser durablement la dépense publique, sinon, cela se solde par plus de dette. Ce financement sera garanti par trois volets d'action. d'abord, je le rappelle, nous allons continuer à nous attaquer aux inefficacités de l'action publique, notamment à tous les opérateurs de l'État dont le fonctionnement et les résultats

le choix d'une politique de l'offre comme politique économique de notre pays. Je le maintiens, parce que je considère que la faiblesse française vient du manque de richesses que nous créons, de la faiblesse de notre compétitivité, d'un outil de production qui doit innover et se robotiser davantage, et que c'est comme cela que l'on améliorera la prospérité de nos compatriotes et des territoires. L'élément clé structurant de notre politique économique restera donc bien l'amélioration de l'offre française : offre de formations, offre de qualifications, offre de produits. La cohérence, cela consiste à dire que le travail doit payer ! Je l'ai dit une centaine de fois à cette tribune et je le répéterai autant de fois que nécessaire : si nous voulons que plus de Français travaillent, il faut que le travail paye davantage. La baisse de l'impôt sur le revenu que le Président de la République a décidée